des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » (et articles 57 et 57 ).

près de 60 % des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » sont consacrés à l'enseignement supérieur. Au préalable, je souligne que les crédits de la mission inscrits dans le budget triennal pour les années 2018 à 2020 progressent moins rapidement que progressent moins rapidement que l'ensemble des dépenses du budget général. Je m'interroge sur cette absence de priorité, sachant que le niveau élevé et croissant des charges à payer de cette mission, depuis 2010, me conduit déjà à douter de la soutenabilité budgétaire de la mission Les crédits du bloc « enseignement supérieur » se caractérisent par une certaine rigidité. En effet, près de 80 % de cette dépense sont constitués des subventions versées aux opérateurs pour charges de service public. Je centrerai donc mon propos sur plusieurs éléments saillants, sur lesquels je souhaite, madame la ministre, appeler votre attention. Le premier point porte sur le plan Étudiants, présenté le 30 octobre dernier. Ce plan traduit une certaine ambition, dont nous vous félicitons ; un montant d'un milliard d'euros devrait ainsi accompagner sa mise en oeuvre durant le quinquennat.

Sans doute, madame la ministre, pourrez-vous nous préciser comment le Gouvernement entend réussir la rentrée 2018-2019. Au-delà de l'accompagnement financier, seule la mise en place d'une professionnalisation de l'orientation, avec un module de plusieurs semaines, permettra de couronner cette réforme de succès. Le deuxième point porte sur la situation budgétaire de certaines universités, qui se servent des attributions d'emplois comme variable d'ajustement pour équilibrer leurs budgets. Plus que jamais, il me paraît urgent que des mesures de rattrapage soient engagées pour les universités sous-dotées. Au reste, cette question se pose dans un contexte particulier. D'abord, les universités sont très inquiètes quant à la remise en cause des fonds de la taxe d'apprentissage et de leur accès à cette taxe. Ensuite, une nouvelle expérimentation de dévolution immobilière sera conduite l'an prochain. Or aucune dotation initiale n'est prévue. Je soutiens la reprise de la dévolution immobilière, gage de l'autonomie des universités, mais il importe de ne pas précipiter le mouvement sans s'assurer que les universités concernées sont effectivement en mesure d'entretenir leur parc. S'agissant des ressources des universités, je considère que les frais d'inscription pourraient être sensiblement relevés, en particulier pour les étudiants étrangers. Il est éclairant de constater que les droits de scolarité ne représentent qu'une part marginale des ressources des universités- moins de 3 %. %. Un relèvement de ces droits permettrait d'améliorer qualitativement l'accueil des étudiants, donc notre attractivité pour faire venir les meilleurs étudiants du monde entier. Le troisième point porte sur les établissements d'enseignement supérieur privé. Je reviendrai sur leur situation financière fragilisée lors de la présentation de l'amendement adopté par la commission des finances. Je souhaiterais toutefois, madame la ministre, que vous nous précisiez comment le Gouvernement compte assurer l'accompagnement de ces établissements. le Gouvernement s'était engagé à clarifier leur situation à travers la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ou EESPIG.

donc à une impasse. Le quatrième point porte sur les crédits destinés à la vie universitaire, le programme 231. Ces crédits paraissent stables par rapport à 2017. Je relève cependant que cette stabilité repose, en réalité, sur la diminution des crédits finançant l'aide à la recherche du premier emploi. Derrière cette stabilité en trompe-l'oeil, les crédits du programme 231 se caractérisent par un fort dynamisme, porté principalement par les facteurs de hausse continue de l'enveloppe dévolue aux bourses. Dans un contexte budgétaire contraint, il importe plus que jamais de s'interroger sur le dynamisme des dépenses. À cet égard, une réflexion sur le contrôle des bourses et de l'assiduité des étudiants devrait être conduite. Je me permets, madame la ministre, de vous signaler les recommandations que j'ai formulées à l'occasion d'un rapport d'information en 2016 sur ce sujet. Elles restent d'actualité et offrent des solutions afin de concilier l'utilité de ce soutien à la poursuite des études et le nécessaire contrôle qui doit les régir. Avant de laisser mon collègue vous livrer son analyse des crédits consacrés à la recherche, je soulignerai le rôle de la recherche universitaire. Près de 4 milliards d'euros lui sont destinés. L'enjeu crucial pour améliorer l'efficacité de cette recherche est d'agir sur le transfert de ses résultats, afin de mieux valoriser les efforts en la matière. C'est tout le sens du travail que j'ai conduit cette année sur les sociétés d'accélération du transfert de technologies, les SATT. J'espère, madame la ministre, que cette étude inspirera votre action, afin de renforcer l'efficacité de l'action des SATT et de parvenir à une à une meilleure valorisation de la recherche universitaire. Avant de conclure, madame la ministre, je veux souligner l'enjeu crucial de la réforme que vous souhaitez engager pour mieux réussir l'orientation et la répartition des étudiants à leur entrée à l'université. l'université. Il y va de l'avenir de nos jeunes, à qui l'on doit arrêter de mentir en les laissant s'entasser dans des filières sans avenir. Il y va aussi d'une meilleure utilisation de l'argent public, donc d'une amélioration des performances de notre enseignement supérieur.

De fait, il était temps que la recherche soit considérée comme un budget prioritaire, au même titre que ceux de la sécurité, de la justice ou de l'éducation, car elle constitue la dépense d'avenir par excellence. Le montant total des crédits alloués aux programmes qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire les programmes 172, « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » et 193, « Recherche spatiale

troisième fait saillant dans les programmes du ministère de la recherche est l'effort budgétaire très important qui sera consenti en 2018 en faveur des très grandes infrastructures de recherche et des organisations internationales

supérieur et de la recherche, verront, pour la plupart, leurs moyens stagner, voire diminuer en 2018. On note deux exceptions à cette tendance morose : le programme 142, Enseignement supérieur et recherche agricoles », qui verra ses crédits augmenter de 2 %, afin notamment de répondre aux besoins des filières agricoles en cadres de haut niveau, le programme 190, « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables », qui bénéficiera de la budgétisation des crédits de recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile qui figuraient, jusqu'en 2016, par les deux premiers programmes d'investissement d'avenir, pour un montant de 135 millions d'euros en autorisations d'engagement. Le fait que l'État apporte de nouveau une aide précieuse à un secteur décisif pour l'avenir de notre industrie, après le « trou d'air » de 2017- si vous me permettez ce jeu de mots -, constitue une excellente nouvelle.

avait montré que la baisse drastique des crédits de l'ANR survenue au début du quinquennat précédent avait eu des conséquences catastrophiques, avec un taux de succès atteignant difficilement 11 % en 2015. Le précédent gouvernement avait fait un effort. On constate, cette année, un effort chiffré qui ne qui ne peut qu'aller dans le sens du renforcement de l'ANR. C'est une bonne chose. Peut-on pour autant considérer que l'objectif que s'est fixé le nouveau Président de la République, à savoir redonner à l'ANR des moyens dignes de ceux de ses homologues étrangers, est atteint ?

En ce qui concerne les financements européens, les premiers chiffres du programme-cadre « Horizon 2020 » pour la recherche en Europe tendent à montrer que le recul de la France en matière de recherche au niveau européen s'amplifie. Si l'Allemagne et la Grande-Bretagne obtiennent traditionnellement plus de financements européens que notre pays, la France est désormais rattrapée par les Pays-Bas et par l'Espagne. Notre pays gagnerait donc

madame la ministre, mes chers collègues, je salue le Gouvernement pour l'effort qu'il consent en faveur de la recherche dans ce budget. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre commission s'est prononcée en faveur de l'adoption des crédits de la mission. Il conviendra cependant de maintenir la hausse des crédits de l'Agence nationale de la recherche dans les futurs budgets du quinquennat,

au vu des avancées de SpaceX, Ariane 6 sera-t-elle suffisamment compétitive pour garantir à l'Europe un accès indépendant à l'espace ? A-t-on pris conscience qu'il est crucial que nos entreprises se saisissent des opportunités économiques de Galileo et de Copernicus ?

Ne devrait-on pas rechercher une plus grande cohérence des structures d'avenir en vue de valoriser la recherche et d'accroître la recherche partenariale ?

d'une société par actions simplifiées, dotée d'un capital de 100 millions d'euros, réparti à parité entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Active depuis 2011, France Brevets est la seule structure publique dédiée à l'investissement dans les brevets en Europe. Elle acquiert des droits sur des brevets en vue de les regrouper en grappes, puis de les licencier, avec pour objectifs de protéger l'innovation française à l'échelon international et de permettre aux entreprises françaises souhaitant utiliser une technologie brevetée de le faire à conditions tarifaires raisonnables. Six ans après sa création, France Brevets doit toujours faire ses preuves. Si son activité est utile, elle s'est surtout développée au gré des opportunités et a donné lieu à des réalisations relativement limitées au regard des objectifs initiaux, alors que ses résultats financiers apparaissent nuancés. La société s'est récemment dotée d'un nouveau plan d'affaires, qui procède à des ajustements bienvenus. Mais, à terme, il faudra procéder à une évaluation indépendante et exhaustive, afin de s'assurer de la valeur ajoutée effective de France Brevets, qui, à ce stade, ne me paraît pas encore totalement démontrée.

madame la ministre, mes chers collègues, en dépit de contraintes budgétaires fortes, le projet de loi de finances pour 2018 témoigne de l'importance qu'attache le Gouvernement à la recherche et à l'innovation, que ce soit à travers l'augmentation des crédits de l'Agence nationale de la recherche ou l'arrêt d'une pratique qui consistait à sous-estimer systématiquement les contributions de la France aux organisations internationales de recherche. C'est la raison pour laquelle la commission de la culture a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Néanmoins, au-delà du budget de la recherche et de l'innovation, il me semble indispensable, surtout en début de quinquennat, de poser la question suivante : quelle recherche veut-on ? Et pour quelle France ? En effet, si notre pays veut rester compétitif, il devra investir massivement dans la recherche et l'enseignement supérieur pour faire de l'innovation le moteur de la croissance économique. Comme l'a dit précédemment mon collègue Jean-François Rapin, avec une dépense de recherche et développement de la France représentant 2,24 % du PIB, notre pays n'a jamais atteint l'objectif de la stratégie de Lisbonne de 2000, qui fixait ce taux à 3 PIB.Les moyens pour y parvenir sont connus : investir davantage dans la recherche publique, mais également encourager le développement de la recherche privée. Soyons honnêtes : jusqu'à présent, aucun gouvernement, toutes majorités confondues, n'y est parvenu. Au cours de la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron s'y est engagé. Nous observerons donc avec attention l'action de l'actuel Gouvernement et ses résultats dans ce domaine. D'ores et déjà, une piste devrait être privilégiée : le renforcement des Instituts Carnot, qui assurent avec efficacité le lien entre recherche et innovation et incitent les entreprises, notamment les PME, à investir dans la recherche. Une autre action doit être menée en parallèle : la définition de priorités claires en matière de recherche. C'est ce qui explique le succès de l'Espagne et du Royaume-Uni dans le cadre des appels à projets européens ou encore le rayonnement de la recherche du Royaume-Uni et des Pays-Bas au niveau international, alors même que ces pays investissent proportionnellement moins d'argent dans la recherche que notre propre pays. C'est un chantier délicat, mais indispensable, auquel le Gouvernement semble vouloir s'attaquer. Nous verrons si, au-delà du constat partagé, les politiques mises en oeuvre seront utiles pour notre pays. Les opérateurs de recherche ont également besoin d'une meilleure visibilité financière à moyen terme pour mener une recherche de qualité. Tel devrait être le rôle des contrats d'objectif et de performance signés entre les organismes de recherche et l'État, avec la mise en place d'une véritable contractualisation des objectifs et des moyens entre l'opérateur de recherche et son ministère de tutelle. Enfin, l'État doit financer les actions qu'il lance. À cet égard, je rappelle que l'INSERM a été chargé par l'ancien gouvernement de plusieurs projets, tels que le lancement du consortium REACTing pour coordonner la recherche en cas d'émergence infectieuse, le pilotage du plan France Médecine Génomique 2025 ou encore la mise en place d'une cohorte dans le cadre du plan de lutte contre la maladie de Lyme- pour ne citer que ces trois exemples. Ces programmes ont été annoncés à grand renfort de communication, mais leur financement n'a pas été assuré et a dû être pris en charge par l'INSERM à travers le redéploiement de ses propres ressources. Cela a été valable pour d'autres organismes de recherche, comme le CNRS. Les arbitrages pour 2018 n'ont pas encore été rendus, mais il serait très regrettable que l'État ne respecte pas ses engagements.

je dois reconnaître, madame la ministre, que la « première mouture » de ce budget, celle qui a été examinée par le Conseil des ministres du 27 septembre dernier, m'avait déçu.

J'espère que vous poursuivrez dans cette voie lors des prochains budgets. Je demeurais néanmoins inquiet, car rien n'était prévu, à ce moment, pour financer l'augmentation des effectifs dans l'enseignement supérieur, ni le scandale de l'échec en licence, alors que, chaque année, nous accueillons 30 000 étudiants supplémentaires dans notre enseignement supérieur, orientés par défaut vers l'université, où seulement un étudiant sur trois termine sa licence en trois ans, ce qui est une honte pour notre pays et sa jeunesse. Mais, du fait de votre parcours professionnel, vous le savez tout autant

Les crédits de cette mission ont donc été abondés de 15 millions d'euros supplémentaires. C'est peu, mais ces crédits seront complétés par des financements sur projets issus des 450 millions d'euros annoncés dans le cadre du Grand plan d'investissement prévu sur la durée du quinquennat. Vous le savez, je soutiens l'ambition de votre réforme, tout particulièrement votre volonté d'améliorer la réussite étudiante en premier cycle, sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années et sur lequel j'ai plusieurs fois eu l'occasion d'interpeller vos prédécesseurs. je serai très vigilant sur les modalités que vous nous proposerez dans le cadre du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, que le Sénat examinera au début de l'année prochaine. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, madame la ministre : si, dans un an, le nouveau dispositif continue de dysfonctionner, nous ne pourrons plus dire : « C'est la faute d'APB » ... Et la récente réforme de l'entrée en master a montré combien les fausses bonnes idées- je pense à ce fameux « droit à la poursuite d'études », que nous n'avions pas véritablement plébiscité au Sénat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il me revient de vous présenter l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur les crédits du programme 190, consacré à la recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. Ces crédits soutiennent les actions de sept opérateurs, compétents dans des secteurs très différents. Les travaux de recherche menés par ces établissements sont essentiels pour répondre aux défis environnementaux de la France et pour réussir notre transition écologique. Ils permettent d'éclairer les décideurs publics lors de l'élaboration de politiques nouvelles, dans des domaines caractérisés par une évolution permanente des connaissances et des techniques. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une légère hausse du total des crédits de ce programme, avec 1,73 milliard d'euros en crédits de paiement et 1,76 milliard d'euros en autorisations d'engagement. Nous avons relevé que les dotations prévues pour les sept opérateurs sont globalement préservées. À cette stabilité d'ensemble s'ajoute un effort spécifique en faveur de la recherche aéronautique, qui vise à prendre la suite de ressources précédemment apportées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir. Si notre commission s'est majoritairement félicitée de la stabilité des crédits en 2018, plusieurs de ses membres ont appelé de leurs voeux, au-delà d'une préservation de l'existant, une revalorisation plus significative de ces derniers, déterminants pour aborder le futur de notre énergie et de nos mobilités. Notre commission a relevé et approuve deux orientations qui guident de plus en plus les activités des organismes soutenus par le programme. Premièrement, nous avons salué les efforts de coopération et de mutualisation entrepris par les différents établissements, efforts qui contribuent à un enrichissement mutuel de leurs travaux, mais aussi à une optimisation des dépenses publiques. Par ces processus de réorganisation, ces organismes s'attachent à établir des priorités dans leurs activités de recherche, ce qui est une démarche très positive, qu'il faut renforcer à l'avenir. Deuxièmement, nous nous sommes félicités des nombreux partenariats établis par ces opérateurs avec la société civile. Ce souci d'ouverture vise à mieux identifier les attentes sociétales, à y répondre plus efficacement, donc,, à améliorer la pertinence et la légitimité de la recherche publique. Une telle approche permet également de développer la coopération entre ces établissements et le secteur industriel, donnant ainsi des perspectives d'application plus directe aux travaux de recherche. Pour conclure, madame la ministre, notre commission considère qu'un engagement financier de l'État à un niveau élevé est indispensable pour maintenir à un degré d'excellence les capacités publiques de recherche dans le domaine du développement durable. Au vu de la stabilité des crédits pour 2018, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Mes chers de ces crédits. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote.

pour 2013 et pour 2017. Préserver les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce n'est pas seulement un arbitrage financier, madame la ministre. C'est un pari en faveur de l'avenir et de l'innovation. Les 718 millions d'euros de crédits supplémentaires de la mission inscrits au PLF pour 2018 sont ainsi massivement dirigés vers les programmes de la recherche. Avec un budget global de 15 milliards d'euros, la recherche fait, certes, partie des « petits » postes de dépenses de l'État, mais ses moyens restent sous-dimensionnés par rapport aux potentialités de ce secteur et, surtout, vous en conviendrez, par rapport aux enjeux considérables qu'il représente pour l'avenir. concerne l'enseignement supérieur, l'augmentation rapide du nombre d'étudiants fragilise l'équilibre financier de la mission, qui stagne à 13,4 milliards d'euros pour les formations et à 2,7 milliards d'euros pour la vie étudiante. Le système craque et risque d'exploser Si nous saluons l'effort public supplémentaire en faveur de cette mission, force est de reconnaître que ses crédits sont insuffisants. Le comité pour la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur estimait ainsi qu'un effort d'un milliard d'euros supplémentaires était nécessaire jusqu'en 2020, pour tenir compte des évolutions démographiques. d'octobre 2017, le Premier ministre a présenté des pistes pour adapter l'enseignement supérieur français à ces nouveaux défis. Pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires, le plan Étudiants va dans le bon sens. La suppression du tirage au sort est une décision salutaire, qui met fin à une situation absurde et injuste. Des mesures énergiques doivent être prises en complément pour accompagner la population étudiante, qui connaît

Le Gouvernement nous promet d'y consacrer un milliard d'euros sur cinq ans, dont 450 millions d'euros au titre du Grand plan d'investissement et 500 millions d'euros dans les budgets successifs du ministère d'ici à 2022. C'est un geste courageux pour nous sortir de l'impasse dans laquelle nous étions placés depuis de nombreuses années. Il Il faudra aussi, comme l'a souligné Colette Mélot au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, que l'enseignement supérieur se marie davantage avec la formation professionnelle pour que les universités travaillent sérieusement sur la question des débouchés professionnels. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Cour des comptes nous interpelle sur la sous-budgétisation de notre contribution aux organismes scientifiques internationaux et aux grandes infrastructures de recherche.

Ce coup de pouce financier est un bon signe, mais les opérateurs de recherche français et étrangers ne peuvent plus se suffit des seules subventions publiques. Il faut, et je crois que cette position fera consensus dans cet hémicycle, améliorer notre visibilité à moyen terme et établir un contrat de confiance sur plusieurs années avec les acteurs de la recherche. Le temps de la recherche scientifique n'est pas toujours celui de l'équilibre budgétaire. Vous avez, madame la ministre, évoqué l'importance d'une visibilité à cinq ans. Nous vous suivons bien entendu dans cette démarche.

comme le Président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, et, d'autre part, que les pouvoirs publics doivent accompagner davantage les opérateurs de recherche dans les candidatures aux appels à projets nationaux et internationaux, notamment en termes de complémentarité des aides.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la démocratisation de l'accès à la connaissance constitue un enjeu fondamental pour permettre à tous nos concitoyens de s'adapter aux évolutions de la société ou, tout simplement, de s'épanouir. La mission « Recherche et enseignement supérieur » doit donc traduire en permanence la place centrale de ces deux politiques publiques pour notre pays. Les crédits de la mission, qui s'élèvent environ à 28 milliards d'euros pour l'année 2018-s'y 2018-s'y ajoutent des crédits prévus par le troisième programme d'investissements d'avenir -, ne sont pas affectés par les efforts budgétaires visant à réduire les dépenses publiques. Pour autant, ils ne répondent pas aux difficultés rencontrées sur le terrain. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, l'urgence est manifeste, comme pourraient en témoigner nos collègues de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication qui, chaque année, mettent en garde le Gouvernement sur la nécessité d'anticiper l'arrivée massive de nouveaux étudiants.

qu'ils ont accumulées tout le long de leur scolarité et de les préparer à leur vie professionnelle, le tout dans un contexte de contraintes financières fortes, sans leur donner les moyens qui auraient dû accompagner le passage l'autonomie. Dix ans après l'adoption de la loi Pécresse, le problème n'est pas résolu. L'affaire du tirage au sort à l'entrée des filières dites « sous tension » est symptomatique de l'absence de prise en considération des difficultés vécues au sein des universités. À la dégradation de leurs conditions de travail, s'est ajoutée la gestion d'un nombre croissant d'étudiants, alors que les capacités d'accueil n'ont pas été renforcées. Je tiens à le préciser, car les filières sous tension ne sont pas uniquement la résultante du déficit d'orientation des élèves- plus de 169 licences Madame la ministre, nous nous réjouissons de la fin de ce tirage au sort qui entrait en complète contradiction avec les principes les plus fondamentaux de notre pays et qui décourageait des vocations dès les premiers pas de nos jeunes dans l'enseignement supérieur. Le plan Étudiants, que vous avez annoncé le 30 octobre dernier, substitue à la sélection arbitraire l'ouverture de nouvelles places dans les filières en tension tout au long du quinquennat. Nous veillerons à ce que cette décision se traduise dans les faits.

et de parcours de formation personnalisés prévus par le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants sont bienvenus. Encore faudra-t-il disposer des moyens suffisants.

La contrainte budgétaire qui continue de peser sur les opérateurs de recherche avec la progression du glissement vieillesse technicité, ou GVT, demeure inquiétante. Les crédits accordés dans le domaine de l'énergie, du développement et de la mobilité durable sont en deçà des besoins. l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, sont en hausse de 32,7 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 133,9 millions d'euros en crédits de paiement, ce qui permettra d'améliorer le taux de sélectivité des projets de recherche. Sans entrer dans le débat sur la pertinence des appels à projets, il est indispensable d'encourager nos chercheurs, qui s'investissent bien souvent sans disposer d'aucune visibilité sur les financements qu'ils pourront obtenir. Enfin, le crédit d'impôt recherche, qui représente une dépense fiscale de 5,8 milliards d'euros, mériterait d'être mieux évalué. Si nous comprenons qu'il a pour objectif d'inciter les entreprises à investir dans la recherche, cette générosité doit s'appuyer sur d'autres leviers, à commencer par une meilleure coopération entre recherche publique et recherche privée. Pour conclure, je saluerai bien évidemment les efforts du Gouvernement pour parvenir à la présentation d'un budget sincère.

la réussite de chaque étudiant dans le supérieur, le développement de l'autonomie des universités et le soutien à la vie étudiante. C'est aussi un choix de transformation et de responsabilité face à la réalité démographique qui n'a pas été appréhendée dans le passé. Je rappelle que 90 000 bacheliers se sont retrouvés, cet été, sans affectation dans un établissement du supérieur. Ce budget s'élève pour 2018 à un peu plus de 16 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 205,6 millions d'euros par rapport à 2017. Nous le savons tous, les investissements dans la recherche, c'est-à-dire en capital humain, ont un effet direct sur la croissance et l'économie françaises. Le projet de loi de finances pour 2018 assume pleinement un renforcement du soutien à la recherche, dont

de l'enseignement supérieur, la mission que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une stratégie plus large. Je pense au projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, présenté voilà deux semaines. Prises ensemble, ces mesures répondent aux défis de l'université : accompagner et favoriser la réussite de chaque étudiant en tenant compte de ses compétences et de ses désirs. Le système actuel est à bout de souffle. Nous ne pouvions plus accepter un taux d'échec aussi important en licence. Nous n'avions plus le droit de fermer pudiquement les yeux sur la précarité de plus en plus forte des étudiants. Nous ne pouvions plus tolérer cette mascarade du tirage au sort. La réforme transformera notre modèle d'orientation, d'accueil et d'accompagnement pour rendre les affectations des bacheliers plus justes et plus efficaces. Ainsi, les crédits demandés pour l'enseignement supérieur augmentent, en 2018, de plus de 200 millions d'euros, conformément à l'engagement de la majorité en faveur de la jeunesse et de l'accès aux études pour tous. Cette hausse permettra de fluidifier les parcours, d'enrichir et de mieux cibler les filières universitaires de premier cycle, particulièrement celles qui sont Elle financera notamment l'extension en année pleine des 1 000 créations d'emplois de la rentrée qui répond au défi de l'augmentation de la démographie étudiante. la hausse de 59 millions d'euros de l'enveloppe consacrée à l'immobilier permettra de financer les projets de réhabilitation des établissements, dans le cadre de contrats de plan État-régions, et la poursuite de l'opération Campus, Campus, qui vise à soutenir le niveau de vie des étudiants en leur rendant 100 millions d'euros de pouvoir d'achat dès 2018. Les aides aux étudiants bénéficieront à près de 15 000 étudiants boursiers supplémentaires en 2018. En effet, les droits d'inscription à l'université et le prix du ticket universitaire ont été gelés à la rentrée 2017, afin de maintenir le pouvoir d'achat des étudiants et de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Face à un sujet aussi crucial pour l'avenir de notre jeunesse et de notre pays, nous nous devons d'adopter une approche pragmatique et raisonnée. Certes, malgré les progrès significatifs réalisés par ce budget, beaucoup reste à faire. Il faudra toujours mettre en adéquation les budgets avec les besoins en postes, l'évolution des filières avec les résultats économiques, la recherche et l'innovation au service du développement de la Nation. Parce que la recherche et l'enseignement supérieur ne sont pas une île, ils doivent s'adapter aux réalités du terrain et à l'évolution de la société et du monde, voire les devancer. Tel est notre objectif.

Pour conclure, madame la ministre, je tiens à saluer votre vision pour l'enseignement supérieur et la recherche. Une vision qui permettra à chacun, quelle que soit son origine sociale, d'exprimer ses talents.

l'examen de la proposition de budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur » intervient vers la fin du débat budgétaire. Nous allons donc apprécier votre intervention à l'aune de celles de vos collègues qui vous ont précédée à cette tribune. Le novice que je suis en cette matière est surpris de découvrir les capacités miraculeuses de cet hémicycle. En effet, alors que M. Darmanin, votre grand argentier, a déclaré que, pour la première fois depuis des années, son gouvernement avait eu le courage « d'inverser la courbe de la dépense publique la plupart de vos collègues nous ont expliqué que leur budget avait été épargné ... Entre le vote des recettes et la discussion des dépenses, environ 7 milliards d'euros d'économies ont disparu. Cet hémicycle a donc la faculté de transformer les « moins » en « plus » ! Dans cette logique, madame la ministre, vous allez donc nous expliquer que votre budget est un budget de transformation

votera contre ! En effet, nous pensons que votre projet de budget se situe dans la lignée de ceux des précédents gouvernements et qu'il consacre l'abandon par la France de la stratégie européenne, dite « de Lisbonne », dont l'objectif était de promouvoir une économie de la connaissance. Alors que nombre de nos partenaires européens ont augmenté, parfois dans des proportions importantes, la part des dépenses publiques destinées à l'enseignement supérieur et à la recherche, la place de la France reste médiocre. Elle a même reculé dans certains domaines. Ainsi, la part des dépenses des établissements d'enseignement supérieur dans le PIB est inférieure à la moyenne de l'OCDE. Plus grave encore, la dépense annuelle par étudiant est en baisse continue depuis 2009. Loin de vos déclarations et de l'annonce d'un plan massif en faveur de l'université, la dure réalité des chiffres de votre budget fait apparaître une baisse, en euros constants, des dotations des établissements universitaires. Plus grave encore, aucune création de postes n'est prévue. Non seulement les universités ne seront pas davantage aidées pour faire face à l'afflux de 35 000 étudiants supplémentaires, mais encore aucun moyen supplémentaire ne leur est octroyé pour mettre en oeuvre les dispositifs imposés par la réforme de l'accès à l'université dont nous aurons à débattre prochainement. Pour bien apprécier l'extrême gravité de la situation, j'aimerais rappeler que des experts de tous bords estiment qu'il faudrait

aux dépens d'opérateurs historiques qui auront à subir, comme tous les ans depuis trop longtemps, de nouvelles réductions de moyens et de postes. Cet acharnement confine à l'absurdité quand il s'agit de l'Institut de recherche pour le développement, dont le budget baisse de plus de plus de 1,5 %, alors qu'il joue un rôle essentiel dans l'action de la France à l'étranger, c'est-à-dire l'un des objectifs prioritaires du Gouvernement. Par ailleurs, je suis très inquiet de la situation très dégradée de l'emploi public dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les suppressions de postes de chercheurs, l'absence de recrutement nouveau, la baisse des postes ouverts au concours du CAPES et la dégradation des conditions financières et matérielles des agents dissuadent de plus en plus les étudiants de se tourner vers toutes ses professions. Cette crise continue des vocations se traduit par une baisse du nombre des titulaires d'un doctorat, ce qui est très inquiétant pour l'avenir de notre recherche. Une autre politique est possible, pas en Utopie, mais dans l'Europe d'aujourd'hui Depuis des années, un dogme bien ancré dans les esprits impose de considérer la dépense publique comme un mal qu'il faudrait combattre. Il y aurait, comme pour le cholestérol, une « bonne dépense », qui serait privée, et une « mauvaise dépense », qui serait publique. comme le mauvais cholestérol, conduirait à la sclérose- je vous rappelle certains propos sur la graisse du mammouth ... Partant de ce principe, il suffirait donc de transférer de l'argent public des opérateurs de l'État vers la recherche privée pour dynamiser tout le système. L'examen des évolutions de notre recherche depuis dix ans montre, sans conteste, que cette stratégie a échoué. Nous avons affaibli notre recherche publique sans favoriser la recherche privée, bien au contraire. Notre voisin, la Belgique, a mis en oeuvre une stratégie inverse avec une éclatante réussite, puisqu'elle est devant nous dans le classement des pays affectant la plus grande part de leur PIB aux dépenses totales de recherche et développement. Autrement dit, l'investissement massif dans la recherche publique a eu un effet d'entraînement très efficace sur la recherche privée. Cet effet de levier a été observé non seulement en Belgique, mais aussi dans tous les pays où des politiques similaires ont été engagées. Alors, madame la ministre, abandonnez vos dogmes, soyez pragmatique et investissez largement dans la recherche publique. Ce sera bénéfique non seulement à notre économie, mais aussi à notre jeunesse, qui a tant besoin que la science et la connaissance redeviennent un projet de vie. Vous aviez

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne m'étendrai pas longuement sur les grandes masses budgétaires de la présente mission. Elles ont déjà été très bien présentées par nos rapporteurs, dont je salue l'excellent travail. raison de son ampleur budgétaire, la mission « Recherche et enseignement supérieur » n'est pas anodine : avec 26,7 milliards d'euros de crédits de paiement, elle constitue le troisième poste budgétaire de la Nation après l'enseignement scolaire et la défense. Et encore faut-il, pour comprendre l'ampleur de l'effort réalisé, prendre également en compte les 6,5 milliards de dépenses fiscales rattachées au crédit d'impôt recherche et les crédits du plan d'investissement d'avenir. Il faut le dire, parce que c'est encourageant : la France investit dans son avenir.

nos rapporteurs, la hausse concerne prioritairement le financement de la recherche. Au sein de ce programme, nous nous réjouissons que les crédits d'intervention de l'ANR continuent leur progression. De même, nous saluons la prise en compte des critiques faites par la Cour des comptes

À court terme, ce financement semble donc assuré. Nous serons extrêmement vigilants, pour que cette annonce se concrétise bien dans le temps par des inscriptions budgétaires correspondantes. Enfin, à l'instar du rapporteur, nous saluons la compensation intégrale du GVT en 2018 dans les budgets des établissements. Ces points de satisfaction n'occultent pas les aspects plus problématiques du présent budget. La situation financière de l'enseignement supérieur privé, en hausse cette année, n'en demeure pas moins préoccupante, l'engagement de l'État ayant baissé de 17 % au cours du précédent quinquennat. De même, on ne peut que s'inquiéter du fait que rien ne soit prévu dans le présent budget pour compenser aux établissements les effets induits de la hausse de la CSG. Nous déplorons également l'absence de dotation d'accompagnement des prochaines dévolutions de patrimoines

des enjeux de la présente mission. Où en est l'université ? Pour répondre à cette question, deux indicateurs méritent de retenir notre attention : d'une part, la France est en queue de peloton dans l'OCDE en termes de dépenses d'enseignement supérieur rapportées au nombre d'étudiants d'autre part, nos établissements ne brillent pas particulièrement dans le classement de Shanghai. Nous le savons, pour que l'enseignement supérieur français demeure compétitif à l'échelle mondiale, il doit se réformer. Le système, si français, des grandes écoles est une bizarrerie dont le corollaire est malheureusement la relégation des universités à un rang subalterne. Il nous faut réussir le rapprochement des grandes écoles et des universités. universités. Nous y engageons-nous vraiment ? Tant que nous n'oserons pas affirmer que la faculté peut être sélective, ce ne sera pas le cas. Tant que nous n'aurons pas remplacé le baccalauréat par une transition plus harmonieuse entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, ce ne sera pas le cas. Tant que nous n'aurons pas enclenché une dynamique pour enfin rapprocher la formation supérieure initiale de l'entreprise, ce ne sera pas le cas. Enfin, tant que nous n'aurons pas pensé l'orientation au lycée bien avant l'année de terminale, ce ne sera pas le cas.

d'un côté, elle affirmait le principe de la sélection à l'entrée du master, mais, de l'autre, elle garantissait un droit à la poursuite d'études qui, malheureusement, vient en pratique alimenter les statistiques de l'échec universitaire.

du groupe Les Républicains préconisent leur revalorisation, en contrepartie de la mise en place d'un système de bourses sur critères sociaux. Je ne sais si c'est la bonne solution, mais cette proposition a le mérite d'ouvrir la réflexion. Les mêmes remarques peuvent être faites en matière de recherche. Nous le savons, la recherche d'aujourd'hui fait le monde de demain. Or le monde demain sera bouleversé par les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Nous pouvons aussi espérer qu'il soit durable. est de taille, car si nous ne réussissons pas ces révolutions, demain, nous n'existerons tout simplement plus. Ces trois axes constituent-ils effectivement les priorités définies par l'État qui se voudrait stratège en matière de recherche ? ne permet de l'affirmer. Au contraire, faute de déterminer et de hiérarchiser des objectifs précis, notre recherche risque de se diluer dans le saupoudrage. Comme pour l'enseignement supérieur, des choix clairs et courageux doivent être faits. Le groupe et courageux doivent être faits. Le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour saluer la confiance retrouvée dans la recherche et l'enseignement supérieur. La civilisation industrielle a fait place à la civilisation de l'innovation et du savoir. L'État doit saisir cette réalité. Dans cette nouvelle civilisation, la richesse ne vient plus des matières premières ou des sources d'énergie. Elle vient plus que jamais de l'homme, de sa créativité.

madame la ministre, mes chers collègues, « la jeunesse n'est qu'un mot », disait Bourdieu. Nous nous accorderons tous en tout cas à dire qu'elle est une chance. D'abord, parce qu'elle est extrêmement diverse : ses origines multiples, qu'elles soient sociales, culturelles ou géographiques, sont autant d'ouvertures au monde, de projets en devenir foisonnants, de lendemains prometteurs qui ne ressembleront pas aux constructions d'hier. Ensuite, elle reste, dans son ensemble, profondément volontariste et lucide. Malgré certains discours ambiants, où ne jaillissent que nostalgie et angoisses quant à l'avenir, elle résiste, elle s'adapte et plonge dans le présent ainsi que dans le futur, cette « parcelle plus sensible de l'instant », comme l'écrivait Paul Valéry. Valéry. Si 78 % des jeunes sont aujourd'hui optimistes quant à leur devenir, ils sont en revanche majoritairement pessimistes sur les sujets qui touchent le monde. Ils ont conscience des problèmes actuels. D'ailleurs, nombre d'entre eux y font face ; ils acceptent le monde tel qu'il est et sont prêts à l'affronter. S'il y a tant d'initiatives de la part de notre jeunesse, que ce soit dans les domaines de l'entreprise, des arts, du sport, de l'environnement ou de l'engagement, c'est grâce à ce réalisme et à cet optimisme de la volonté, qui nourrissent ce désir de transformer le monde, de l'améliorer, de mieux vivre tout simplement. Albert Camus écrivait que « chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde ». Si une partie de la jeunesse est en capacité de le faire, une autre n'a même pas la possibilité de s'y projeter. Au fond, ce n'est pas une affaire d'ancien ou de nouveau monde. C'est plutôt une affaire de sens. Quel sens donner au monde ? Quel sens donner à ses propres engagements ? Je crois que les jeunes générations ont une conscience particulièrement aigüe et se posent constamment ces questions. Probablement est-ce cette quête permanente de sens qui les conduit à imaginer, concevoir et entreprendre tant d'initiatives, sans être tétanisés d'emblée par le risque d'échec. C'est pourquoi nous avons une responsabilité collective envers la jeunesse, et je dirai même envers toute la jeunesse : celle de lui offrir les meilleures conditions pour apprendre, comprendre et réaliser ses projets. En un peu moins de quarante ans, la France a réussi son pari d'amener nombre d'élèves d'une même classe d'âge au baccalauréat, le taux de réussite passant de 64 % en 1980 à presque 90

est sa capacité à accueillir, à former convenablement tous les jeunes qui désirent légitimement poursuivre leurs études et à les insérer dans la société. Il faut le rappeler, le droit d'accès à l'enseignement supérieur demeure un principe cardinal, qui est à réaffirmer.

nous fait comprendre qu'il n'est plus possible de poursuivre dans cette voie. Madame la ministre, vous avez présenté la réforme que vous souhaitez mettre en oeuvre afin de favoriser la réussite étudiante. Je ne m'y appesantirai pas, dans la mesure où nous débattrons prochainement, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, de ce projet de loi dans l'hémicycle. En revanche, j'attire votre attention sur un constat partagé par nombre d'acteurs universitaires, et en particulier le président de la Conférence des présidents d'université, selon lequel « le projet de loi de finances pour 2018 ne peut être, en l'état, considéré à la hauteur des enjeux par les universités. Certes, le Gouvernement effectue un effort en augmentant les crédits affectés à l'enseignement supérieur d'environ 1,5 %, soit 190 millions environ, complétés, à l'Assemblée nationale, par l'ouverture de crédits, à hauteur de 15,5 millions d'euros, en faveur des formations supérieures et de la recherche universitaire. Néanmoins, cette hausse est malheureusement en deçà des 250 millions d'euros qui seraient nécessaires en vue d'accueillir décemment de 30 000 à 40 000 nouveaux étudiants.

Autrement dit, il se révèle primordial que les moyens alloués à l'université continuent de croître intensément pendant cette période. Je doute que le milliard d'euros annoncé pour financer votre réforme, sur l'ensemble du quinquennat, soit suffisant ... Si tel n'est pas le cas, la responsabilité collective que j'évoquais en introduction, et qui a pour finalité de créer un environnement propice au succès de nos étudiants, commandera de trouver des financements supplémentaires. Quoi qu'il en soit, la réforme et l'accroissement des effectifs ne doivent pas peser sur le budget de fonctionnement des universités, déjà notoirement mis à mal.

les inégalités sont toujours patentes. En effet, si le taux d'élèves boursiers atteint 40 % en première année dans certaines universités, il n'est plus que de 10 % à 12 % en master. Cette statistique n'est pas si surprenante : elle n'est que la continuité de l'étude PISA, qui conclut que notre système éducatif, sans être déficient, est le plus inégalitaire parmi ceux de l'OCDE. Une politique éducative de rééquilibrage, qui part du primaire jusqu'au supérieur, est donc impérieuse. En corollaire, le plan pour la vie étudiante que vous avez décliné, madame la ministre, a le mérite de s'attaquer à certaines barrières susceptibles d'empêcher les étudiants de suivre le cursus voulu le logement, la santé, la complexité à concilier études et emploi rémunéré, enfin la mobilité, facteur vraisemblablement le plus discriminant et le plus violent. violent. Quant à la recherche, elle constitue bien sûr les promesses de demain. Depuis les travaux de l'économiste Paul Romer, l'importance de la recherche pour la croissance, le développement et le rayonnement d'un pays est démontrée. À l'heure où l'économie et la société sont de plus en plus régies par la connaissance, ainsi que par l'exploitation de données, la recherche a un rôle encore plus fondamental.

Par exemple, il est intéressant de citer les polémiques incessantes autour du réchauffement climatique ou de l'efficacité des vaccins. Ainsi la stratégie nationale de CSTI, portée avec volontarisme par notre ancienne collègue Dominique Gillot, pour objet d'améliorer l'accessibilité et la diffusion de cette culture. Elle cible la population française dans son ensemble, mais se focalise principalement sur un public prioritaire, les jeunes de 3 ans à 20 ans.

tous les secteurs d'activité, il pourrait s'avérer pertinent de coordonner les efforts de recherche à l'échelle européenne, afin d'éviter que des pays n'investissent massivement dans les mêmes directions et n'aboutissent aux mêmes découvertes. Piloter les spécialisations aurait la vertu de faire émerger des champions européens par domaine d'activité. Madame la ministre, vous avez conforté, voire fait progresser, deux budgets essentiels qui représentent l'avenir de la Nation. Si nous soutenons votre ambition pour l'enseignement supérieur, nous restons néanmoins perplexes quant à l'adéquation des moyens avec cette

le groupe Les Républicains se félicite que les crédits consacrés à la recherche soient globalement en hausse de 4,6 %, comme l'ont rappelé les rapporteurs. Cet effort était indispensable, car la recherche a clairement été la mal-aimée du précédent gouvernement, dans lequel l'enseignement supérieur et la recherche ne disposait même plus d'un ministère à part entière autant, suffira-t-il à faire revenir nos nombreux chercheurs installés à l'étranger et à retenir ceux qui envisagent de partir vers des pays où l'instabilité en matière de financements et, surtout, l'énergie qu'ils doivent consacrer pour les décrocher est moindre Je le souhaite, mais nos chercheurs auront besoin de plusieurs années pour être enfin rassurés sur la place que la France entend réellement leur donner. Je ne citerai que le cas emblématique d'Emmanuelle Charpentier. Formée en France, elle a découvert avec l'Américaine Jennifer Doudna le système CRISPR-Cas9, utilisé maintenant dans les laboratoires du monde entier, qui révolutionne l'ingénierie du génome humain, animal et végétal. Après la Suède et les États-Unis, c'est à l'Institut Max Planck qu'elle travaille, n'ayant pas pensé un seul instant revenir en France. Tous ces pays ont sans doute la chance de ne pas bénéficier du filtre de l'ANR,

Autant que la faiblesse des crédits qui lui étaient affectés, c'est la procédure de sélection des appels à projets-moins de 12 % d'entre eux étaient retenus -qui a fini de décourager les équipes de chercheurs et provoqué des démissions, et même une fronde des prix Nobel.

de l'ESA. La double présidence, assumée par Jean-Yves Le Gall, est de nature à rassurer tous ceux qui, comme moi, soutiennent la recherche et l'industrie spatiale française, cette dernière ne pouvant se développer que dans le cadre européen. Depuis la conférence de Naples, en 2012, l'industrie spatiale européenne a su se structurer, avec un maître d'oeuvre principal pour les lanceurs, Airbus Group, et trois maîtres d'oeuvre concurrents pour les satellites, Airbus, Thales et Le programme des lanceurs spatiaux et le centre spatial guyanais, confortés dans ce budget, doivent permettre d'assurer à l'Europe son indispensable autonomie d'accès à l'espace. J'espère que les 133 millions d'euros prévus en 2018 pour les systèmes spatiaux de télécommunications et Galileo seront suffisants. Comme notre rapporteur Daniel Dubois, je trouve que l'ESA a été bien longue à faire la promotion du GPS européen,

Si, par le passé, je me suis interrogée sur l'opportunité de continuer à financer la station spatiale internationale, la belle opération de promotion de l'espace menée à l'occasion de la mission de Thomas Pesquet me fait dire qu'elle vaut bien 240 millions d'euros. Je profite

oui ! Mon dernier point portera sur la recherche industrielle. Mes propos seront à la fois plus critiques et plus interrogatifs, car, en ce domaine, l'érosion du soutien que l'on constate depuis plusieurs années n'est pas freinée dans ce projet de loi de finances.

aux crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », il ressort un sentiment assez général, partagé par la plupart des groupes politiques de notre assemblée, de bienveillance globale. Il me semble en effet que nous sommes nombreux sur ces travées à considérer que ce budget a été construit sur des bases de sincérité, avec la volonté de répondre aux importants enjeux liés à cette mission. En hausse de 2,7 % sur les autorisations d'engagement, ce premier budget du quinquennat vise d'abord à digérer les dernières mesures salariales prises l'an dernier, il est vrai en pleine période électorale. Il envoie aussi un signal positif aux élèves et étudiants de notre pays, au moment même où vous présentez un plan Étudiants, sur lequel je reviendrai. Toutefois, cette bienveillance s'accompagne d'une vigilance. d'abord souligner l'augmentation constante des effectifs dans l'enseignement supérieur. Avec les pics démographiques des années 2000 et 2001, et de façon encore plus accentuée entre 2005 et 2014, il s'agit surtout de prendre en compte l'évolution positive du nombre de bacheliers et du taux de poursuite dans l'enseignement supérieur. Pour ne donner qu'un chiffre, la projection du ministère fait apparaître 361 000 inscriptions supplémentaires à la rentrée 2025, comparativement à 2015. est indiqué dans le rapport pour avis de Jacques Grosperrin, c'est le signe d'un dynamisme évident et aussi la promesse d'une réussite pour notre pays. Chacun le sait ici, gouverner, c'est prévoir. Il est donc légitime de s'interroger sur les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour répondre à cette augmentation. Par ailleurs, chacun le sait également, la répartition des étudiants par filière est très inégale. Elle ne répond pas toujours à des besoins réels en termes de débouchés et conduit à des tensions récurrentes. Nous touchons là au délicat sujet de l'orientation, à propos duquel je valide pleinement à la fois les diagnostics et les préconisations de l'excellent rapport réalisé l'an dernier par Guy-Dominique Kennel. Madame la ministre, je partage les objectifs d'accompagnement et de meilleure orientation des élèves, notamment pour pallier le taux d'échec important en licence, constaté de manière si régulière depuis plusieurs décennies. Le processus d'orientation s'inscrit dans un temps long. Il doit évidemment tenir compte des aspirations de chaque élève, mais nécessite aussi une analyse de ses aptitudes à suivre tel ou tel cursus. lors, permettez-moi de douter de l'efficacité de certaines mesures du plan Étudiants, prises dans la précipitation, notamment la désignation d'un second professeur principal dans chaque classe de terminale, dans un délai très contraint, alors même que, pour cette mission chronophage et peu valorisée, on peine à trouver suffisamment de volontaires.

Quand allons-nous cesser de faire faire aux professeurs tout et n'importe quoi, sans formation préalable ? Pourquoi oublier délibérément dans ce dispositif les conseillers d'orientation-psychologues ? Cela traduit-il la volonté de faire disparaître cette profession ? Voilà beaucoup d'interrogations auxquelles le plan Étudiants ne répond pas. Une orientation réfléchie doit aussi se traduire par une affectation cohérente. Quoi qu'on en dise, la procédure APB, admission post-bac, a rendu dans ce domaine les services attendus lors de sa mise en place. Elle est victime aujourd'hui d'effectifs devenus trop importants. Il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. À titre personnel, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'ancien monde n'a que de mauvais côtés ! Très bien ! Une chose est sûre : personne ne pouvait accepter que perdure le tirage au sort effectué cet été encore pour attribuer des places dans quelques filières sous tension. Comment expliquer en effet à un bachelier ayant obtenu une mention « très bien » que sa candidature n'a pas été retenue, au bénéfice d'un camarade moins méritant ? Sur la forme, madame la ministre, vous aurez sans doute contenté un certain nombre d'internautes en leur laissant choisir le nom - ParcourSup - de la prochaine procédure d'admission dans le supérieur. Au-delà Au-delà de cet exercice participatif et, disons-le, quelque peu accessoire, le nouveau système proposé, pour ce que l'on en sait, c'est-à-dire pas grand-chose, inquiète les différentes parties concernées, alors que le calendrier s'annonce des plus serrés. Il inquiète les élèves de terminale, qui n'ont que très peu d'informations sur les modalités de formulation des voeux, sur les conséquences de l'absence de classement de ces voeux et, sur la décision des établissements d'accueil. Il inquiète également les professeurs et proviseurs de lycées, qui auront la lourde tâche, dans quelques semaines, d'expliquer le fonctionnement de la nouvelle plateforme aux élèves et à leurs parents. Il inquiète enfin les établissements de l'enseignement supérieur, qui peinent parfois à recruter suffisamment d'étudiants. Je pense ici aux classes préparatoires, que je connais bien, puisque, il y a encore deux mois, j'enseignais au sein de l'une d'elles. En remplaçant l'algorithme de tri d'APB par un algorithme de temps, certaines de ces classes, parmi les moins prestigieuses, devront attendre fébrilement les réponses positives des futurs bacheliers, sans aucune visibilité sur leurs effectifs à la rentrée. J'y vois une menace sur le maintien de cette spécificité française, qui conditionne les parcours d'excellence que nombre de pays nous envient. Sur le fond, la procédure ne sera pleinement efficiente que si les places offertes dans l'enseignement supérieur correspondent à un réel besoin pour notre pays. On peut évidemment concevoir que le souhait de chaque candidat soit une composante essentielle, mais le rôle des gouvernants est d'avoir une vision globale et de fixer le cap. Il faut donc en finir avec le sacro-saint droit à l'université pour tous. Bien sûr, il y a des parcours scolaires atypiques ; bien sûr, il faut laisser la place au droit à l'erreur d'aiguillage. Mais cessons de nier l'évidence des inscriptions fantaisistes au sein de nos universités ! Vous avez fait un pas en suggérant- que dis-je, en susurrant ! -que des attendus pourraient être exigibles à l'entrée à l'université. La sémantique a été soignée pour éviter même le terme de prérequis je considère que la sélection n'est pas une vilenie, que cela constitue même un service à rendre à tous ceux qui subissent deux ou trois années d'échec.

Une autre mesure régulièrement repoussée, parfois pour de bonnes raisons, souvent par dogmatisme, consisterait à revaloriser les droits d'inscription. Là aussi, j'ai noté sur ce sujet récurrent une certaine convergence au sein de la commission des finances. Il y va de la compétitivité de nos universités, qui peinent aujourd'hui à rivaliser sur le plan mondial. L'autonomie ne suffit pas, il faut permettre aux universités d'avoir les moyens de leurs ambitions. d'inscription devrait, bien sûr, s'accompagner d'une augmentation compensatrice des bourses sur critères sociaux pour les familles modestes. Elle ne devra pas être un prétexte, pour l'État, à se désengager. Peut-être pourriez-vous, madame la ministre, clarifier la position du Gouvernement sur ce point ? Enfin, le Gouvernement a annoncé une réforme du baccalauréat. Je forme le voeu que celle-ci soit ambitieuse, pour redonner de la valeur à ce premier diplôme de l'enseignement supérieur. L'un de mes collègues du lycée où j'enseignais avait ce bon mot pour décrire la situation actuelle de cette évaluation : « Il ne faut jamais sous-estimer la capacité du bac à se faire avoir ». Au-delà de la boutade, cette formule traduit le mal-être profond En diluant les enseignements, en multipliant les options obligatoires ou facultatives, on a donné la possibilité d'obtenir le baccalauréat sans valider ses connaissances dans les matières fondamentales. Pis, aucun contrôle d'assiduité ne vient réellement faire obstacle à certains élèves, qui, en dépit d'absences injustifiées répétées, peuvent se présenter aux épreuves et obtenir ce sésame pour l'enseignement supérieur. Un enseignement de qualité ne peut être dispensé que par des professeurs motivés et convaincus de l'utilité de leurs cours. J'espère que ce modeste témoignage pourra trouver un écho dans la réflexion qui sera menée pour réformer cette institution. Puissions-nous éviter, cette fois, un nivellement par le bas le bas ! Madame la ministre, réformer l'enseignement supérieur pour permettre une meilleure orientation et une meilleure réussite des étudiants est une belle ambition, que nous partageons. Un grand chantier a débuté avec le plan Étudiants, pour lequel vous avez augmenté les crédits de la MIRES, la mission Pour l'exercice budgétaire à venir et les suivants, nous serons vigilants et veillerons à ce que leur utilisation réponde de manière effective aux enjeux majeurs auxquels nous devons répondre, dans l'intérêt de notre jeunesse. La parole

La première de mes priorités a été de rétablir la sincérité de la programmation budgétaire. Comme nombre de nos concitoyens, j'ai pris toute la mesure des questions soulevées par la loi de finances pour 2017 lors de la publication du rapport de la Cour des comptes. C'était malheureusement trop tard pour reconnaître au Sénat le mérite d'avoir mis en évidence la sincérité parfois discutable de ce texte, mais assez tôt pour prolonger cette réflexion sur nos finances publiques et en tirer toutes les leçons. Le budget de la MIRES qui vous est proposé pour 2018 est le produit de ce travail, lequel nous a conduits à apporter des réponses à ces deux questions : comment rétablir la sincérité des crédits inscrits dans le budget ? Comment traduire sur le plan budgétaire la politique du Gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche ? Vous le savez, le soutien à nos établissements d'enseignement supérieur et à nos laboratoires fait partie des priorités cardinales du Gouvernement, qui a placé au coeur de son action la construction de notre avenir commun. C'est pourquoi ce projet de budget prévoit une forte hausse des crédits relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ces crédits progressent de plus de 700 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, en s'établissant à 24,5 milliards d'euros. La MIRES, dans son ensemble, disposera de 27,7 milliards d'euros, hors intérêts de la dette. C'est donc le troisième poste budgétaire de notre nation. C'est un effort considérable qui est ainsi fait au service de la préparation de notre avenir, de celui de notre jeunesse au travers de notre enseignement supérieur, mais aussi de celui du pays tout entier, qui se nourrit des progrès de la recherche et de leur diffusion rapide, par l'enseignement et l'innovation. C'est également un budget stratégique, qui finance l'effort de la Nation en matière spatiale et contribue ainsi au rayonnement international de notre pays. Nos concitoyens sont sensibles à cet effort et aux défis posés par la recherche scientifique. L'aventure scientifique continue de susciter leur intérêt, que ce soit dans le domaine spatial ou, plus récemment, dans les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle.

et entrer dans la compétition internationale. Nous devons permettre à nos laboratoires de se projeter dans un temps long et dans un monde de plus en plus concurrentiel. C'est pourquoi nous avons choisi d'augmenter de plus de 500 millions d'euros les crédits consacrés à la recherche,

Par ailleurs, nous voulons redonner de l'oxygène à nos chercheurs, qui souffrent depuis des années de financements insuffisants et des querelles doctrinaires opposant les partisans de la recherche sur projets et les défenseurs du financement récurrent. À ce débat, j'ai souhaité apporter une réponse claire : nous avons besoin des deux ! Une recherche financée intégralement sur projets serait perpétuellement fragile et soumise à tous les aléas de la conjoncture économique et scientifique des laboratoires financés sur des seuls crédits de base ne pourraient permettre l'émergence des idées neuves. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen de l'amendement de M. Ouzoulias. Sans préempter cette discussion, ma volonté, ainsi que celle du Gouvernement, est de financer ce qui fonctionne, donc de réaffirmer le soutien à la recherche dans son ensemble, 140 millions d'euros Le budget de l'ANR sera ainsi porté à 750 millions d'euros. Et, afin d'améliorer le taux de sélection des appels à projets, sa capacité d'engagements sera portée à 706 millions d'euros, afin d'amorcer le le retour vers un taux de sélectivité qui ne sera plus totalement contre-productif. Par ailleurs, les instituts Carnot verront leurs crédits augmenter de 5 millions d'euros ; ils ont fait la preuve de leur efficacité pour établir des partenariats performants, équilibrés et fluides avec le monde économique. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises : c'est un modèle de financement de la recherche intéressant, qui mériterait d'être diffusé. Toutefois, cela ne signifie pas que nous délaissons les crédits de base. Bien au contraire, nous avons pris une décision inédite dans la période récente : nous avons choisi de dégager quelque 25 millions d'euros en direction des laboratoires, afin d'augmenter les crédits de base. En effet, chacun connaît la réalité, dans les universités comme dans les organismes les financements récurrents avaient tellement baissé que nos unités de recherche n'avaient plus les moyens de conduire un projet scientifique propre au long cours. Ces 25 millions d'euros constituent une première respiration, qui, là aussi, devra être amplifiée, mais qui représente une rupture avec ce qui était devenu une forme de dogme : la réduction permanente des crédits de base au profit de la recherche sur projets. En parallèle, nous travaillons à réduire les fragilités financières structurelles du secteur, en rétablissant au bon niveau les financements destinés aux très grandes infrastructures de recherche, qui sont l'un des fers de lance de notre science à l'échelle internationale. Là encore, trop longtemps, la programmation d'ensemble, scientifique et budgétaire, de ces projets n'a pas été suffisante, et ce sont les organismes de recherche qui étaient contraints de prendre en charge sur leurs budgets le poids issu du dérapage desdits projets.

en étroite collaboration avec le ministère de l'action et des comptes publics, pour prévoir une augmentation des crédits : sur le long terme, ce sont près de 314 millions d'euros supplémentaires qui serviront à donner un surcroît de sincérité aux crédits budgétaires des organismes internationaux. Concernant l'enseignement supérieur, vous le savez, 2018 sera une année tout à fait particulière, puisque nous mettrons en oeuvre la réforme de l'orientation et de la réussite à l'université, qui constitue la colonne vertébrale du plan Étudiants que j'ai présenté, avec le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, le 30 octobre dernier. Ce plan Étudiants, le Gouvernement l'a construit afin de répondre à une double urgence : d'une part, le recours au tirage au sort pour l'accès à l'enseignement supérieur, qui a concerné en 2017 plus de 66 500 étudiants la lutte contre l'échec en premier cycle, auquel nous nous sommes finalement lentement habitués- j'en veux pour preuve les documents budgétaires eux-mêmes, au sein desquels le taux de réussite en licence en trois ans figure parmi les indicateurs de performance, avec une cible, à l'horizon 2020, de 30 % ... Aujourd'hui, nous sommes à 27 % de réussite. C'est de cette situation que nous devons sortir, en accompagnant nos étudiants vers la réussite, car ce taux d'échec est la chose la plus injuste socialement À cet égard, j'adresse mes remerciements anticipés à M. Grosperrin, qui sera le rapporteur du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, et je salue Guy-Dominique Kennel et Catherine Procaccia, dont les travaux, ces dernières années, ont inspiré largement les pages de ce texte qui sera examiné par le Sénat en février prochain.

Étant attentive aux travaux conduits notamment par le Sénat, permettez-moi de vous apporter d'emblée quelques garanties, afin de répondre à ceux qui ont pu, très récemment, mettre en doute la parole du Gouvernement devant la Haute Assemblée. Ainsi, je rappelle que le Premier ministre a annoncé il y a cinq semaines un effort supplémentaire de plus d'un milliard d'euros, par rapport à un budget en croissance de plus de 700 millions d'euros. Cet effort supplémentaire se décompose ainsi : 450 millions d'euros, d'abord, au titre du Grand plan d'investissement, afin de financer la transformation pédagogique du premier cycle de licence et de construire de nouveaux cursus personnalisés. Un premier appel à projets sur les nouveaux cursus universitaires a déjà ses lauréats et mobilise plus de 130 millions d'euros ; le second appel à projets vient d'être lancé

500 millions d'euros de crédits budgétaires supplémentaires afin de créer des places dans les filières de premier cycle en tension et dans les formations courtes professionnalisantes, notamment en BTS et en DUT. Cet effort permettra de créer des postes, de financer des heures d'enseignement supplémentaires et de reconnaître l'engagement pédagogique des enseignants et des enseignants-chercheurs. Cet engagement s'est traduit dès cette année par une série d'amendements

100 millions d'euros supplémentaires seront rendus aux étudiants en pouvoir d'achat grâce à la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante dès 2018. Jusqu'alors, les étudiants devaient payer 217 euros en plus chaque année au titre de l'assurance maladie, alors même qu'ils n'avaient, dans leur grande majorité, aucun revenu. C'était une anomalie ; elle sera corrigée, et les étudiants, tous les étudiants, y compris les étudiants internationaux bien sûr, bénéficieront d'une couverture gratuite et d'une qualité de service et d'accès aux soins nettement améliorée. Le plan Étudiants n'épuise pas, tant s'en faut, la question du financement de notre enseignement supérieur, qui appelle quelques développements, afin que vous soient présentés les objectifs du Gouvernement en la matière pour l'année à venir. Tout d'abord, j'ai souhaité nous sortir collectivement d'une mauvaise habitude, celle de dissimuler sous des budgets en hausse apparente diverses impasses budgétaires, qui venaient ronger peu à peu les marges de manoeuvre réelles. C'était particulièrement crucial pour l'enseignement supérieur, car, depuis plusieurs années, nos universités et nos grandes écoles doivent résoudre une quadrature impossible : d'un côté, la démographie étudiante est en hausse, on le sait depuis environ de l'autre, les charges ne cessent d'augmenter, sous l'effet notamment du glissement vieillesse technicité, qui n'a pas été financé au cours des dernières années. La conséquence de cette quadrature a été simple : là où les lois de finances affichaient des créations de postes, la réalité, dans les universités, était celle de l'utilisation des crédits supplémentaires pour couvrir la progression permanente des charges. Tout à fait ! C'est avec cette logique délétère que nous avons rompu cette année, en remettant enfin à niveau les budgets de nos universités et en finançant le GVT. En tant qu'ancienne présidente d'université, je mesure parfaitement l'ampleur de cette petite révolution. Cet effort inédit portera les moyens de l'enseignement supérieur à plus de 13,4 milliards d'euros sont 194 millions d'euros de plus par rapport à 2017. Et si l'on s'attache aux crédits qui seront effectivement disponibles pour les établissements, ce sont même 234 millions d'euros de plus qui seront notifiés aux universités et aux grandes écoles grâce à la baisse du taux de mise en réserve. Enfin, afin de financer les projets de réhabilitation de l'immobilier des universités dans le cadre des contrats de plan État région, ainsi que la poursuite de l'opération Campus, l'enveloppe consacrée pour 2018 à l'immobilier s'élèvera à 343 millions d'euros, soit une augmentation de presque 60 millions d'euros. maintenant, pour répondre aux différentes questions qui ont été posées au cours de cette discussion générale. Je commencerai par la question du plan Étudiants. De façon générale, je souhaite l'articuler avec deux autres réformes qui ont commencé la réforme du baccalauréat, portée par Jean-Michel Blanquer, qui, bien sûr, a été complètement associé à l'élaboration du plan Étudiants, et la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de la formation continue et de la formation tout au long de la vie, portée par Muriel Pénicaud, réforme à laquelle, bien sûr, nous sommes associés, Jean-Michel Blanquer et moi-même. Il faut bien le comprendre, ce que nous souhaitons, c'est à la fois repenser l'orientation dès la fin du collège ou le début du lycée

l'importance de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur ! Sur ce sujet, monsieur Adnot, je souhaite vous rassurer : la taxe d'apprentissage continuera à financer les formations de l'enseignement supérieur.

Je vous confirme, monsieur Ouzoulias, que l'acharnement confine parfois à l'absurdité. Il ne faut pas opposer la recherche de base et la recherche sur projets. Et il était très important de redonner aussi de la respiration à la recherche sur projets, tout simplement parce qu'elle permet à de jeunes équipes et à de jeunes chercheurs de s'émanciper, de porter un projet, donc de poser les bases et la fondation d'une future unité mixte de recherche. Il est donc absolument essentiel que nous soyons en capacité de faire émerger, par la recherche sur projets, nos équipes de recherche d'excellence de demain. Le taux de financement de l'ANR, avec une sélectivité extrêmement forte,

financements extrabudgétaires qu'elle contrôle, de financer un certain nombre de plans. En effet, madame Darcos, vous avez raison, de nombreux plans nationaux ont été annoncés

de lancer des plans nationaux. Le premier, sur le climat, a été engagé et confié au CNRS ; il y en aura un sur l'intelligence artificielle, confié à l'INRIA,

Nous comptons agir de deux façons différentes. Tout d'abord, je participe extrêmement activement à l'ensemble des commissions qui se déroulent à l'échelon européen. Évidemment, si l'on est absent de ces commissions, on a un peu de mal à préparer

plan relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, la plateforme sera présentée avant les vacances de Noël. Je souhaite rassurer tout le monde : je n'ai jamais dit

nous oblige aujourd'hui à changer de système, et nous ne pouvons pas conserver un algorithme entièrement automatisé. C'est pourquoi nous en avons imaginé un autre, qui est en simulation, qui fonctionne, et que nous aurons le plaisir de présenter avant les vacances de Noël. Il est de notre responsabilité à tous, nous, adultes, de rassurer les lycéens sur le fait que

Accompagner la réussite, reconnaître les talents, quels qu'ils soient, soutenir l'optimisme de notre jeunesse, c'est selon moi la meilleure protection de la démocratie. Nous allons

Lorsqu'il s'agit des collectivités territoriales, nous sommes tous d'accord pour limiter, voire réduire, le « mille-feuille territorial ». Dans le domaine de la recherche, en revanche, nous assistons à un bourgeonnement baroque de structures à la fois coûteuses, bureaucratiques et inefficientes. L'Agence nationale de la recherche est l'une de ces Elle est devenue une agence à dire « non », puisque la proportion des projets qu'elle finance n'a cessé de diminuer, pour atteindre un plancher d'environ 10 % ; mais, pour cela, il lui faut de plus en plus de personnels. Ainsi, cas exceptionnel dans le budget de la recherche, elle va bénéficier de trente emplois supplémentaires. collègues, son budget de fonctionnement a été multiplié par dix, le nombre de ses personnels par quatre, mais les fonds qu'elle distribue seulement par un et demi ! Le nombre de chercheurs diminue, mais le nombre de personnels administratifs chargés de gérer leurs demandes, lui, augmente

la langue de la République ... -, a préféré confier la sélection des propositions scientifiques de la communauté internationale aux CRS-

J'ai écouté avec attention votre discours, madame la ministre : vous avez dit vous-même que les grands fonds nationaux que vous alliez lancer allaient être financés par les opérateurs historiques- vous avez cité l'INRIA, le CNRS, etc. Pourquoi ne pas les confier à l'ANR, si vous avez tant confiance en cette agence ? ! Sur le fond, je partage votre sentiment : on ne peut pas opposer la recherche financée par des crédits récurrents et la recherche sur projets. J'ai moi-même fait les deux-

pour les redéployer vers le programme 150. Je rappelle que l'ANR n'a pas pour vocation de porter les grands plans nationaux ; ce sont bien les organismes de recherche qui les portent.

Les chercheurs sont soumis à un régime qui les épuise. Aussi, lorsqu'ils obtiennent un statut, ils ont malheureusement dépensé l'essentiel de leur énergie à courir après les financements. Ce modèle ne fonctionne pas ! Il provoque des drames humains considérables et il est, du point de vue de la recherche, contre-productif.

des étudiants est catastrophique. Un quart d'entre eux bénéficient d'une bourse dont le montant maximal se situe autour de 555 euros, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, et 50 % des étudiants sont salariés. Ce dernier chiffre doit faire réfléchir

à peu près qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Sur leurs conditions d'études, les étudiants expriment de façon quotidienne leur fatigue ; ils nous parlent d'une sorte de combat pour la survie.

puisé dans les crédits dédiés aux établissements privés, qui représentent environ 18 % des étudiants. L'objectif n'est pas de les supprimer- j'ai déjà dit ici que j'étais favorable à la liberté d'enseignement, et même à la libre-pensée ! Toutefois,

Il n'empêche que vous avez raison de dénoncer les inégalités entre les jeunes, car elles existent. À mon sens, la plus criante d'entre elles n'est pas celle qui existe entre le public et le privé,

Monsieur Adnot, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, je n'oppose absolument pas les établissements publics aux établissements privés, surtout lorsqu'il s'agit d'établissements privés d'intérêt général et qui sont donc sans but lucratif.

cette année, 9 nouveaux établissements ont obtenu la qualification, parmi lesquelles 3 écoles d'ingénieurs d'agriculture qui bénéficient d'un contrat avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Les autres sont principalement des écoles de management. Au total, 56 établissements bénéficient donc de la qualification d'EESPIG pour cette année.

Les établissements privés d'enseignement supérieur, à l'image de leurs confrères des premier et second degrés, constituent aujourd'hui des accélérateurs d'inégalités sociales ». Ce n'est pas faux ! Je suis profondément scandalisé de lire

Nous sommes pour la réussite des jeunes enfants. Je prends l'exemple de la Bretagne, où près d'un élève sur deux est scolarisé dans un réseau autre que celui de l'enseignement public,

de ses enfants. Pour ma part, je salue le travail qui est effectué par Mme la ministre et je pense, mes chers collègues, que la plus grande des inégalités est celle qui est règne aujourd'hui à l'université, où on laisse croire à beaucoup de jeunes qu'ils réussiront dans leur parcours universitaire, alors qu'ils n'y ont pas été préparés. Je rappelle que deux étudiants sur trois quittent l'université avant d'avoir obtenu un diplôme et se retrouvent sur une voie d'échec.

En favorisant les échanges avec la communauté scientifique, en opérant un partage des savoirs et en éduquant les publics à une citoyenneté active, elle inscrit la science dans la société. à l'enseignement supérieur et à la recherche a clarifié les rôles entre l'État et les régions. Ces dernières se sont vues transférer la coordination et la mise en cohérence des actions de la CSTI. Les régions ont bien un rôle central dans la nouvelle gouvernance de la CSTI : organisation du réseau des acteurs sur leur territoire, engagement des projets, soutien financier des actions portées dans ce domaine. Pour autant, les crédits nationaux décentralisés, s'ils viennent bien abonder ces financements régionaux, ne le font qu'à hauteur de 4,7 millions d'euros. L'État conserve encore des moyens d'action non négligeables ; il doit rester un acteur incontournable pour donner le goût de la science aux nouvelles générations. Vous pouvez penser que la réussite de la CSTI dans le cadre d'un contexte budgétaire restreint repose davantage sur la rationalisation de la gouvernance que sur une augmentation des moyens. Pour ma part, je ne le crois pas. Il est selon moi nécessaire aujourd'hui de promouvoir auprès des jeunes publics le goût de la science. Il s'agit aussi de résorber l'écart entre l'évolution des sciences et des techniques et la capacité des citoyens à la comprendre pour la maîtriser. Or les avancées scientifiques ont été si importantes ces dernières années que nous avons tout à gagner à ce que chaque citoyen devienne plus savant, donc plus responsable et moins naïf. Comprendre pour mieux faire des choix de société, n'est-ce pas un idéal à poursuivre dans une société avancée ? ? Nous en sommes à un moment crucial, particulièrement en la matière, s'agissant des choix relatifs à l'énergie, l'écologie, etc. Cette question touche également celle des stéréotypes de genre ; il est urgent de développer cette culture afin d'encourager les jeunes filles à se diriger vers les carrières scientifiques et techniques. Pour ces raisons il est nécessaire de donner un nouveau souffle au développement des politiques partenariales : État, collectivités, associations. Au printemps dernier, le Conseil national de culture scientifique, technique et industrielle, présidé par Dominique Gillot, a remis la stratégie nationale de CSTI. L'ambition fixée par cette dernière nécessite un investissement supérieur aux moyens actuels consacrés à la CSTI qui ne peut pas être assuré par les régions seules. C'est pourquoi il est proposé de reprendre la proposition du Conseil national et d'augmenter les crédits d'intervention. Bien évidemment, je ne veux pas porter atteinte au financement de la recherche duale. Je souhaite néanmoins que le Gouvernement se saisisse de ce sujet et que la Haute Assemblée puisse prendre toute sa part à

Je profite de cette intervention pour saluer le travail important réalisé par votre ancienne collègue Dominique Gillot, qui s'est fortement investie. La Nation consacre La Nation consacre déjà 250 millions d'euros spécifiquement à la CSTI : 196 millions d'euros dédiés aux musées et aux établissements publics

Malheureusement, les crédits de la recherche duale sur lesquels vous voulez prendre les finances pour la CSTI ne me permettent pas d'émettre un avis favorable sur cet amendement.